s'apparente donc à une TVA sociale, car elle finance une baisse de charges sociales ; c'est une position connue des centristes. Elle pourrait d'ailleurs tout aussi bien s'appeler « TVA compétitivité », car elle est remboursée à l'exportation et payée à l'importation. Elle fait donc contribuer l'ensemble des entreprises étrangères au financement de notre système de protection sociale, ce qui permet de financer la suppression de la hausse de la CSG.

la baisse de cotisations sociales, mais va directement dans les caisses de l'État. Ces opérations budgétaires entre finances sociales et finances de l'État nous conduisent à en appeler à une réflexion d'ensemble sur l'impôt et sur les prélèvements sociaux. est l'objet de cet amendement. Plusieurs questions méritent d'être posées. Est-il juste que les retraités financent les baisses de cotisations sociales bénéficiant aux actifs ? Est-il juste que tous les Français ne contribuent pas aux finances sociales à concurrence de leurs moyens ?

n'aura aucune compensation. Avouons-le clairement : on cherche à faire payer par une partie des retraités l'augmentation d'un certain nombre de prestations,

je n'y étais pas, pour ma part, hostile -entre les retraités et les actifs. Or une convergence, cela signifie aussi les mêmes conditions pour ce qui concerne les compensations.

Les membres du groupe socialiste et républicain, avec conviction, et unanimement, demandent la suppression de l'alinéa 9 de l'article 7. La solidarité est est exigeante de justice sociale. Aussi, la proposition d'augmentation de la CSG pour les retraités n'est pas, selon nous, acceptable. Elle est même destructrice de notre cohésion sociale quand, dans le même temps,

la compensation de la hausse de la CSG pour l'ensemble des catégories, sauf pour les retraités, au motif que le montant des pensions de retraite a progressé plus rapidement que celui des salaires. Il nous semble tout à fait injuste de considérer que cette évolution due, comme je l'ai expliqué hier, à la plus forte activité des femmes, ferait des retraités des privilégiés par rapport aux salariés.

la fiscalisation des majorations familiales, décidées sous le quinquennat précédent. Cette accumulation de mesures nous semble peu respectueuse du rôle social, je dirais presque sociétal, joué par les retraités, de leur aspiration, qui me semble tout à fait légitime, à vivre le moment de retraite comme un temps plein, un moment d'épanouissement. Nous dénonçons cette politique de stigmatisation à l'égard des retraités, quand 60 % d'entre eux vivent avec une pension proche du seuil de pauvreté, situé à 1 015 euros par mois. Pour la grande majorité d'entre eux, il est même de plus en plus difficile de se soigner. Nous demandons au contraire une revalorisation de toutes les retraites, afin qu'aucune d'entre elles notamment ne soit inférieure au SMIC. Tel est le sens de cet amendement.

M. Daudigny ne l'a pas exprimé, que la hausse de la CSG ne concerne pas les titulaires de pension d'invalidité. En effet, cette hausse ne sera compensée par aucune baisse de cotisation, puisque les pensionnés n'en paient pas. Cela représente une perte nette de pouvoir d'achat de plusieurs centaines d'euros par an. Pire encore, les quelques revalorisations obtenues lors des quatre dernières années seront en fait complètement couvertes

ont été menées par l'Association des paralysés de France. Mais plus encore que la question financière, monsieur le ministre, il s'agit ici d'une question de dignité pour les titulaires de pensions d'invalidité. Exclus malgré eux du travail, ils le sont aussi souvent sur le plan social, quand ils ne sont pas dans une profonde détresse économique. Les personnes invalides comme les personnes handicapées ressentent ces attaques comme autant de relégations. La pension d'invalidité, l'AAH, ne sont pas censées devenir des minima sociaux, et leurs bénéficiaires n'ont rien d'assistés. C'était d'ailleurs l'un des combats que portait très fortement notre ancienne collègue Annie David, que je veux ici saluer et qui a choisi de passer la main.

tend à ce que la contribution des retraités à cette réforme soit non pas supprimée, mais atténuée pour les plus modestes. Celle-ci ne s'appliquerait qu'aux retraités ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 18 500 euros annuels, contre 14 375 euros dans le projet du Gouvernement. Cela permet de sortir de la réforme 10 % de retraités, en préservant leur pouvoir d'achat. Je rappelle, mes chers collègues, que nous parlons ici de retraités ayant des pensions de moins de 1 500 euros. J'ajoute que les effets de seuil seraient limités, par le maintien d'un taux à 6,6 % situé entre le taux réduit de 3,8 % et le taux après réforme de 8,3 %. Enfin, le dispositif prévu assure la transition pour 2018 de la hausse de la CSG avec la mise en oeuvre du dégrèvement en trois ans de la taxe d'habitation.

Cette hausse aura des conséquences diverses sur le pouvoir d'achat des Français. Pour les salariés, elle sera compensée par la baisse des cotisations sociales, laquelle n'interviendra pas de manière totalement concomitante à la hausse de la CSG. En 2018, pendant plusieurs mois, cela risque de faire perdre du pouvoir d'achat aux Français. Pour les fonctionnaires, le Gouvernement annonce une compensation à hauteur de 3 milliards d'euros, qui, pour l'heure, n'a pas fait l'objet d'engagements inscrits au projet de loi de finances. Pour les retraités, la hausse s'appliquera à ceux qui sont actuellement assujettis au taux de 6,3 %. Ainsi, pour une personne seule, cette hausse s'appliquera dès que le revenu fiscal de référence dépasse 14 375 euros, soit 1 289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans, et dès 1 394 euros par mois si elle a plus de 65 ans. Ainsi, un retraité avec 1 400 euros par mois aura à payer en plus 285 euros de CSG. Afin d'obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d'achat des retraités français et l'exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, il est proposé que la hausse de CSG pour les retraités ne s'applique pas pour les montants de retraite inférieurs au coût moyen d'une maison de retraite médicalisée.

verra sa CSG augmenter et les cotisations sociales diminuer- il y a donc un gain de pouvoir d'achat, nous en avons conscience et nous le saluons -et il verra aussi,

Cependant, pour les professionnels de santé libéraux, dont les cotisations maladie et famille sont prises en charge, en totalité ou en partie, par l'assurance maladie, notamment les médecins de secteur 1, la mesure de réduction dégressive des cotisations prévue pour les travailleurs indépendants ne permettra pas de compenser la hausse de CSG, compte tenu de cette prise en charge préexistante. Des avenants conventionnels doivent donc être conclus au plus vite avec les professions concernées, afin de prévoir des mesures de compensation équitables et sans discrimination pour chaque profession de santé.

Monsieur le ministre,

Le projet de loi vise à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles, actuellement fixé à 3,04 %, par un taux progressif s'étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel. la Mutualité sociale agricole, cette mesure a un coût de 120 millions d'euros pour l'agriculture française. Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles. En effet, depuis le 1 janvier 2016, les exploitants agricoles bénéficient d'un taux de cotisation fixe de 3,04 résulte d'un engagement pris par l'État en 2016 en vue, d'une part, de redonner de la compétitivité aux exploitants agricoles français et, d'autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens. Ces engagements s'étaient traduits par la baisse de sept points de la cotisation d'assurance maladie et maternité applicable dès 2016. L'application de la mesure présentée conduirait à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d'un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit 75 % du SMIC. Avec la hausse de la CSG prévue à cet article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d'une compensation intégrale ; ceux qui ont, au contraire, des revenus plus élevés- un peu plus élevés -subiront une perte de 5 points de revenus. Or tout le monde le sait ici, dans leur majorité, les agriculteurs ne roulent pas sur l'or.

et n'a nul besoin d'être davantage maltraitée. Cet amendement, vous l'avez compris, vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d'assurance maladie et maternité. Je crains, monsieur ministre, que nous n'ayons pas mesuré de cette mesure, qui conduirait en effet à ce que seuls les agriculteurs ayant de faibles revenus bénéficient d'une compensation intégrale. On parle là d'un revenu de 13 500 euros par an ! Monsieur le ministre, je vous laisse méditer

Or, dans le projet de loi de finances pour 2018, ces 437 millions d'euros sont supprimés pour être remplacés par 300 millions d'euros de dotation provisionnelle pour dépenses imprévisibles.

problème. On entend partout les cris des agriculteurs, et il ne me semble pas que ce soit le moment d'ajouter encore de la détresse à une détresse déjà largement exprimée. L'amendement n° 410 est présenté par M. Marie.

la cotisation d'assurance maladie et maternité, dès 2016, pour redonner des marges de compétitivité et pour rapprocher les taux de prélèvements sociaux de ceux de nos voisins européens. Le Gouvernement décide de changer la donne et de passer d'un taux de cotisation maladie et maternité de 3,04 % à un taux progressif de 1,5 % à 6,9 %. Au premier abord, cela pourrait paraître séduisant, puisque les plus faibles revenus en seront les principaux bénéficiaires. Cela étant, quand on examine de près les montants des gains en cause, on s'aperçoit que, pour un revenu

On demande donc tout simplement que le taux de 3,04 % soit maintenu et que l'ensemble de la profession agricole puisse en bénéficier. Rappelons au passage qu'un revenu

on peut le constater, depuis un certain temps, le niveau des exportations agroalimentaires françaises n'est pas au beau fixe ; il est plutôt en baisse.

de notre pays et, surtout, à la force de l'agroalimentaire français. Voilà ce que je voulais ajouter aux propos de mes collègues, parce que, derrière cela, il y a des femmes et des hommes et il y a toute la puissance de notre agriculture. C'est un signe de reconnaissance du travail quotidien de celle-ci.

Le Gouvernement a engagé une transformation du régime social des indépendants. Confier la protection sociale des indépendants au régime général suppose d'harmoniser les cotisations et les prestations y afférent. En alignant la protection sociale des agriculteurs sur le régime général, la rédaction actuelle de l'article 7 aurait pour effet de baisser le taux des cotisations jusqu'à 1,5 % pour les exploitations agricoles les plus modestes. En revanche, pour les agriculteurs dont les revenus professionnels sont supérieurs à 20 000 euros, cette harmonisation se traduirait par l'annulation d'une partie de la baisse de charges du taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité de sept points, décidée en 2015. Aussi, pour ces exploitations agricoles, le taux de cotisations pourrait passer de 3,04 % à 6,5 %, selon le montant des revenus professionnels. Il est, par conséquent, proposé de plafonner le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des agriculteurs à 3,04 %, afin que la réforme envisagée par le Gouvernement permette une harmonisation par le haut pour notre agriculture, dont la compétitivité est essentielle, je le rappelle, pour notre pays.

L'instauration d'un système plus progressif n'est pas mise en cause, mais il conviendrait indubitablement de mieux calibrer le dispositif, pour éviter de précariser

l'avis de la commission ? Tout le monde l'aura compris, cet amendement vise à supprimer le principe de la réduction dégressive de la cotisation maladie des exploitants agricoles. Le taux de la réduction est fixé par voie réglementaire. En mars 2016, dans le cadre d'un plan d'urgence pour l'agriculture, le Gouvernement avait baissé uniformément de sept points, sans considération du revenu, le taux de cotisation des exploitants agricoles, qui a ainsi été fixé à 3,04 % pour les années 2016 et 2017. Cette mesure a été financée par le ministère de l'agriculture, pour un montant de 520 millions d'euros. D'après l'étude d'impact, la moitié de cette somme, j'y insiste, a bénéficié aux 15 % des exploitants agricoles dont les revenus sont les plus élevés.

dont nous discutons, il est prévu d'harmoniser le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles avec celui des autres travailleurs indépendants, avec une réduction dégressive allant de 1,5 % à 6,5 %, selon le revenu.

Le dispositif proposé est néanmoins plus ciblé sur les agriculteurs à bas revenus, pour lesquels la cotisation maladie est divisée par deux. Au total, selon les chiffres fournis- peut-être M. le ministre pourra-t-il les confirmer ou les ou les infirmer -, 57 % des exploitants agricoles seraient gagnants avec la mesure proposée. La commission s'est déterminée en essayant de savoir quelle était la mesure la plus juste

aucun agriculteur ne connaîtra une situation stagnante ou défavorable par rapport à l'année 2016. C'est le premier point,

Le rapport de la Cour des comptes a démontré que la dérive budgétaire du ministère de l'agriculture au cours du quinquennat précédent représentait 7 milliards d'euros, et la France est incapable, depuis des années, de se mettre en accord avec la politique européenne. D'où des apurements communautaires qui nous coûtent une fortune.

la Cour des comptes évoque jusqu'à 7 milliards d'euros sous le quinquennat précédent -, alors que tout cet argent pourrait utilement être utilisé pour l'agriculture française. Il n'est donc pas juste et, surtout, il n'est pas raisonnable

les jours ! Les agriculteurs en font tous les jours, l'école en fait tous les jours, les collectivités locales en font tous les jours, la santé en fait tous les jours, les quartiers en font tous les jours, la ruralité en fait tous les jours ... C'est un débat de responsabilités.

largement rappelé, leur vote est une nécessité pour l'ensemble de la profession agricole. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos arguments, mais, quel que

vos commentaires. Je peux moi aussi beaucoup dire sur le précédent gouvernement, mais je crois qu'aujourd'hui les Françaises et les Français attendent autre chose

cette aide était obligatoire tant que la compétitivité n'était pas retrouvée. Mais, aujourd'hui, qui peut dire que la compétitivité des exploitations agricoles françaises sera retrouvée

par les apurements communautaires après de multiples appels et relances de la Commission européenne, c'est parce que l'administration française n'a pas spécialement fait son travail.

Pourtant, pour l'administration française, depuis 1992, cet hectare n'a jamais été le même. Il a fallu faire une déclaration cadastrale en 1992, une déclaration photo un peu plus

non, on offre à l'agriculture française les conditions pour lutter sur la scène européenne. Monsieur le ministre, vous le savez très bien, la seule politique qui existe en matière de formation des prix et des charges est communautaire.

amendement. Il faut tout de même souligner, et c'est un point que personne, y compris M. Le Foll, à l'Assemblée nationale, n'a pu contredire, qu'il s'agissait bien d'une mesure non pérenne.

La première année de la trajectoire budgétaire que nous proposons, cette augmentation de CSG serait compensée par la suppression de la taxe d'habitation. Ne divisons pas

quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des agriculteurs, non pas pour qu'ils se vantent de ce qu'ils font sur le territoire, mais parce qu'ils rencontraient des problèmes de revenus, notamment de RSA. De fait, dans les départements, le nombre d'agriculteurs bénéficiaires du

revenus fonciers et plus-values immobilières s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Ainsi, à titre d'exemple, une vente d'immeuble ou de terrain agricole réalisée en juin 2017 sera taxée à un taux supérieur de 1,7 % au taux connu par le contribuable au moment de la cession. Or une telle rétroactivité aurait pour effet d'appliquer des règles d'imposition autres que celles qui étaient applicables à la date du fait générateur. Elle porterait ainsi atteinte à des situations légalement acquises.

l'avis de la commission ? En l'absence de retenue à la source, le changement des règles fiscales s'applique évidemment aux revenus soumis à l'imposition à l'année n+1. Il en sera de même pour la mise en place du prélèvement forfaitaire unique,

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, un amendement introduit par le Gouvernement est venu modifier la taxation de l'épargne salariale. Il est ainsi prévu que les nouvelles plus-values réalisées par les salariés seront désormais soumises intégralement au dernier taux connu de prélèvements sociaux, et ce dès le 1 janvier 2018. Le régime précédent, dit des « taux historiques », était plus favorable dans la mesure où les plus-values étaient taxées au taux en vigueur au moment de leur constatation. Les épargnants n'avaient donc pas à subir le renchérissement des prélèvements sociaux sur leurs versements passés. Cette mesure prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale alourdira à terme la taxation de l'épargne des salariés. Ce serait un très mauvais signal adressé aux 11 millions de salariés qui détiennent un compte d'épargne salariale, notamment à ceux- les plus modestes -qui ne disposent que de cette seule épargne financière après une vie entière de labeur. Cet alourdissement, même limité, n'incitera pas les épargnants à conserver leur portefeuille de titres sur le long terme, ce qui paraît incohérent avec les réformes engagées par le Gouvernement en faveur de l'épargne longue et avec les annonces

deux mois et demi. Aussi, il est demandé de revenir sur cet objectif et de permettre à l'ensemble des salariés disposant d'un plan d'épargne d'entreprise de continuer à bénéficier du taux historique de leur épargne salariale. Quel

La suppression des taux historiques ne vaut que pour l'avenir. Les prélèvements sociaux sur ce type de revenus sont fixés à 17,5 % depuis 2012.

cet article prévoit que le revenu attaché aux sommes versées dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 1 janvier 2018 ou au cours des cinq premières années suivant un versement, lorsque celui-ci est intervenu entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2017, reste soumis aux taux historiques.

Si les choses restaient en l'état, ces petits exploitants subiraient donc une perte de pouvoir d'achat en 2018, par rapport à 2017, contrairement à l'ensemble des autres actifs du secteur privé. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que le taux de la cotisation applicable en 2018, et fixé par décret, ne puisse excéder le taux applicable en 2017, qui serait diminué de 2,15 points, soit 13,85

est à Mme Catherine Morin-Desailly. Améliorer le pouvoir d'achat des actifs, c'est la raison invoquée par le Gouvernement pour justifier la hausse de 1,7 point de la CSG, rendue nécessaire pour pallier la baisse des cotisations salariales des salariés. Pour les artistes auteurs, cette réforme ne devrait pas se traduire par des gains de pouvoir d'achat. Écrivains, compositeurs, chorégraphes, scénaristes, photographes, plasticiens ne profiteront pas de la baisse des cotisations d'assurance chômage, et pour cause : leurs revenus sont essentiellement ou totalement tirés des droits d'auteur et des ventes d'oeuvres, et les droits d'auteur ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à l'indemnité chômage. Les artistes auteurs vont donc voir leur rémunération diminuer, et c'est là un effort loin d'être insignifiant, compte tenu de la précarité à laquelle cette profession est parfois confrontée. Le Gouvernement avait promis de trouver une solution à l'Assemblée nationale- le débat a été lancé dans cette enceinte -, mais il n'en a rien été. Il est indispensable que la hausse de la CSG puisse, à tout le moins, être compensée pour cette catégorie d'actifs. C'est une question d'équité.

À qui profitera cette mesure ? Aux « artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques », dont il est question à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Pourquoi se contenter de poser un principe ? Tout simplement parce que la loi renvoie à un décret le soin de fixer le taux de la cotisation vieillesse. Par parallélisme des formes, il appartient donc au pouvoir réglementaire de fixer le montant de la réduction octroyée aux artistes auteurs. J'attire néanmoins l'attention du Gouvernement sur la nécessité que la prise en charge soit égale à 0,95 point de cotisation, pour permettre une compensation de la hausse de la CSG pour les artistes auteurs.

madame la sénatrice,

C'est vraiment la concrétisation de la suppression des cotisations, à la faveur d'une fiscalisation la CSG. Monsieur le ministre, vous soutenez cette CSG, son augmentation même, sous prétexte de solidarité intergénérationnelle, voire d'universalité.

Qu'est-ce qu'une cotisation sociale, si ce n'est un salaire différé ? Quoi de plus juste ? Au lieu de la conforter, nous allons le voir tout au long de l'examen de ce texte, vous multipliez les exonérations, notamment patronales. Vous fiscalisez

de santé - par les bénéficiaires eux-mêmes. La fiscalisation du financement de la protection sociale participe directement

des lois de financement de la sécurité sociale pour 2015 et 2016, le Sénat avait décidé de supprimer cet assujettissement.

Si la loi est aujourd'hui discriminatoire, elle est de plus l'expression d'un contresens économique, comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer précédemment. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire

Sénat. Les députés de la majorité précédente n'ont donc pas fait confiance avec constance aux entrepreneurs, surtout aux travailleurs indépendants, qui pourraient, je cite, fictivement « faire passer pour des dividendes la rémunération de leur activité

Le précédent gouvernement a laissé perdurer, à partir de 2013, une situation injuste, puisque les Français établis à l'étranger paient la CSG et la CRDS sans bénéficier des prestations correspondantes, est par ailleurs contraire au droit de l'Union européenne. Pour les Français de l'étranger, la hausse de la CSG et de la CRDS, c'est double imposition et double peine La France a déjà été condamnée en février 2015 dans l'affaire de Ruyter par la Cour de justice de l'Union européenne, suivie quelques mois plus tard par le Conseil d'État. Résultat : l'État a dû rembourser les sommes indûment perçues. suite de la condamnation de la France, le précédent gouvernement avait décidé de modifier le fléchage de la CSG-CRDS, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, en affectant les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine principalement au Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, mais aussi à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. En procédant ainsi à compter du 1 janvier 2016, au détriment de nos compatriotes installés à l'étranger, la France a certainement ouvert la voie à un nouveau contentieux avec la Commission européenne, car le règlement communautaire précise bien que ces règles s'appliquent aussi aux prestations spéciales à caractère non contributif. La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour violation du droit communautaire. Monsieur le ministre, le redressement des finances publiques ne peut pas passer par une fiscalité abusive et contraire au droit européen. Je vous ai d'ailleurs adressé pas plus tard qu'hier un courrier afin de savoir où en est la procédure d'infraction engagée par la Commission européenne contre la France. Notre amendement vise donc non seulement à remédier à une injustice à l'égard des Français de l'étranger, mais aussi à épargner à la France une nouvelle condamnation par les instances communautaires.

Le Gleut, le vote du projet de budget rectificatif de l'été 2012 a introduit l'assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux, ce qui a entraîné une double imposition pour ceux-ci.

Cette décision a été confirmée par le Conseil d'État quelques mois plus tard et a ouvert la voie à de nombreuses réclamations auprès du fisc, dont l'impact budgétaire est évalué à environ 300 millions d'euros pour la seule année 2013, ce qui n'est pas rien. L'État a malheureusement persévéré dans une analyse plus que fragile juridiquement. Le produit de la CSG a été affecté au Fonds de solidarité vieillesse et celle-ci constitue donc, selon l'État, un impôt non contributif, et non pas une cotisation sociale. Outre que cette analyse juridique est d'ores et déjà infirmée par la jurisprudence européenne, le coeur du problème tient au respect du principe constitutionnel d'égalité. Assujettir une personne à un prélèvement social alors qu'elle n'est pas affiliée à un régime obligatoire français, c'est tout d'abord la contraindre à subir une double imposition sociale, en France et dans son pays de résidence, mais également à cotiser sans contrepartie, c'est-à-dire sans bénéficier de prestations. Pour rappel, une procédure d'infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents est toujours en cours. Je crois donc, monsieur le ministre, qu'il est temps de renoncer au prélèvement de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents, sans attendre une nouvelle condamnation de la Cour de justice

en 2013 sur l'assujettissement des Français de l'étranger à la CSG et la CRDS sur leurs revenus du capital ».

qu'il existait une contradiction entre, d'une part, notre droit interne et les décisions du Conseil constitutionnel, qui considérait que la CSG était une imposition de toute nature, et, d'autre part,

Aujourd'hui pèse toujours sur nos finances publiques la menace de nouvelles condamnations,

Il ne s'agit pas ici des conséquences de l'arrêt, comme le disait M. Le Gleut : cet arrêt concernait, je le rappelle, un résident fiscal en France de nationalité néerlandaise, affilié à la sécurité sociale dans son pays d'origine.

FSV. Notre commission n'était pas hostile à ce que ces revenus du patrimoine et des produits de placement, dégagés en France, puissent contribuer au financement des dépenses de solidarité.

Nous avons conscience d'être légèrement à contre-courant des politiques d'exonération et d'exemption de cotisations de sécurité

de mener une politique sociale audacieuse pour répondre aux besoins actuels et futurs, car nombreux sont les défis à relever.

Ce dispositif est complexe, mais pas forcément beaucoup plus que le mécanisme de contribution des entreprises productrices de médicaments. Au travers de cet amendement d'appel, nous entendons inciter le Gouvernement à mettre en place un autre financement de la sécurité sociale, visant à encourager les entreprises vertueuses qui pratiquent une politique salariale et sociale positive, notamment en privilégiant une répartition des richesses favorable

près de 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Au total, près d'un tiers des femmes travaillent à temps partiel. Ce phénomène n'est pas dû au hasard, mais à des discriminations sexistes qui existent dans les sphères privée et publique : en particulier, ce sont très majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants hors temps scolaire. Les ordonnances de M. Macron, dans la droite ligne de la loi éponyme et de la loi El Khomri, vont malheureusement accentuer cette tendance, puisque le plancher minimal de vingt-quatre heures hebdomadaires est totalement dérogatoire. Nous pensons au contraire qu'il est essentiel de mettre fin